La séance est reprise. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Philippe François, qui fut sénateur de la Seine-et-Marne, de 1983 à 2004. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Jean Louis Masson. Madame

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les débats qui ont eu lieu sont tout de même très instructifs.

préservant la région Alsace. Absolument ! Si la voix du Sénat avait été entendue, nous ne serions probablement pas aujourd'hui réunis pour examiner un projet de loi visant à créer une Collectivité européenne d'Alsace.

! Malheureusement, dans de nombreuses régions, on constate plutôt une augmentation des dépenses ! Trois ans après l'entrée en vigueur du texte, je ne suis toujours pas à l'aise avec cette nouvelle région Grand Est, qui est trop vaste et, surtout, dépourvue d'. Tout à fait C'est pour ces raisons que nous souhaitons donner une réalité juridique, législative, à un fort « désir d'Alsace », exprimé par une très large majorité d'Alsaciens, 84 % selon les derniers sondages. désir d'Alsace » a été très bien observé et compris par Mme la ministre, Jacqueline Gourault, que je tiens à remercier de son excellent travail. Ainsi que cela a été rappelé, ce désir aurait pu prendre plusieurs formes. Le Gouvernement a choisi ce qu'on pourrait appeler une fusion de départements améliorée, aboutissant à la création d'une collectivité dénommée « Collectivité européenne d'Alsace Ce choix me conduit à formuler un regret. Je regrette que nous n'ayons pas pu aller plus loin et aboutir à la création d'une collectivité à statut particulier. cela aurait été la meilleure solution. Pour autant, même si j'aurais donc préféré aller plus loin, je reconnais, associant mon collègue Jean-Marie Bockel l'intérêt du compromis auquel nous sommes parvenus avec le Gouvernement. Ce compromis a abouti à la signature à l'hôtel Matignon, le 29 octobre 2018, d'une déclaration commune en faveur de la création d'une Collectivité européenne d'Alsace. J'apporte donc mon soutien au projet de loi qui nous est proposé aujourd'hui. Ce soutien ne m'empêche pas de formuler certaines réserves à l'égard du texte initial déposé sur le bureau du Sénat. Les travaux de la commission des lois ont permis de lever la plupart de ces réserves. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail de notre rapporteur, Agnès Canayer,

évoquer les avancées les plus importantes adoptées par la commission. Le nouvel article 2 prévoit que la Collectivité européenne d'Alsace pourrait à titre expérimental se voir déléguer par la région l'octroi de tout ou partie des aides aux entreprises. Tout département pourrait d'ailleurs demander à bénéficier de la même expérimentation. Après l'adoption d'une disposition similaire dans le cadre de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, adoptée le 13 juin

Sans dessaisir la région, un tel mécanisme permettra d'introduire de la souplesse dans les politiques locales de développement économique. À l'article 3, c'est à juste titre que la commission des lois a attribué le pouvoir de police de la circulation sur les autoroutes non concédées au président de la collectivité. Merci ! Il était effectivement nécessaire de clarifier les règles applicables aux autoroutes transférées. Enfin, il n'était pas souhaitable que les règles relatives à la composition du collège électoral concourant à l'élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin intègrent le champ de l'habilitation prévue à l'article 9. Je me félicite que la commission ait adopté mon amendement sur ce point et que la rapporteur ait introduit, à l'article 8, la répartition des conseillers départementaux et régionaux élus dans la section correspondante entre les collèges appelés à élire les sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

voilà l'intitulé figurant à la fois dans la déclaration commune signée à Matignon le 29 octobre 2018, dans le décret du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin- je précise que c'est la fusion des des deux conseils départementaux, et non des deux départements -et dans le présent projet de loi. Pour un Alsacien comme moi, comment défendre un autre intitulé aujourd'hui ? C'est celui sur lequel est fondé l'accord qui est l'objet même du projet de loi que nous examinons. Contre l'avis du rapporteur, nos collègues du groupe socialiste et républicain ont fait adopter un amendement prévoyant la création d'un « département d'Alsace ». Pour nous, il s'agit d'une remise en cause du projet que nous défendons. Je regrette que cette modification ait été intégrée au texte de la commission, même si je suis si je suis d'accord pour dire que toutes les collectivités françaises ont une mission européenne. Je soutiendrai donc sans réserve les amendements visant à rétablir l'intitulé : « Collectivité européenne d'Alsace Malgré ce dernier aspect, je tiens une fois encore à saluer la qualité du travail réalisé par la commission des lois. À l'exception du nom de la collectivité, le texte qu'elle nous propose aujourd'hui est enrichi, sans que soient remis en cause les équilibres initiaux défendus par le Gouvernement.

La dénomination " Collectivité européenne d'Alsace " a disparu ; vive le département d'Alsace ! » C'est ainsi que pourrait s'intituler la chronique d'une mort annoncée. Non, nous ne voulons pas d'un simple « département d'Alsace », qui ne correspond pas au mandat que les Alsaciens nous ont confié ! Le « désir d'Alsace », porté par les deux présidents des conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, a conduit le Gouvernement à exprimer une volonté d'accompagnement qui nous semblait pourtant claire. Mais était-elle aussi explicite et aussi volontariste ? J'ai encore la faiblesse de le croire. à l'hôtel de Matignon, arraché aux forceps au Gouvernement, a créé la Collectivité européenne d'Alsace, le 29 octobre dernier. Cette collectivité doit être dotée de compétences élargies, de compétences élargies, supradépartementales, dans les domaines dans lesquels l'Alsace excelle ou doit se renforcer, comme la coopération transfrontalière, le tourisme, le bilinguisme ou la mobilité. Fin de l'acte I. Il nous fallait attendre les deux délibérations concordantes des conseils départementaux, puis le décret en Conseil d'État, et enfin le texte de loi ; c'est chose faite. Fin de l'acte II. nous allons écrire ensemble l'acte III d'un événement historique qui pourrait se terminer en drame ou en espoir pour les Alsaciens, les citoyens et les élus, tous unis pour défendre le même objectif. Mais loin de moi une démarche de repli ! Nous voulons assurément que l'expérience alsacienne puisse être transposable, pour ce qui concerne certaines de ses compétences élargies et renforcées, à d'autres territoires. Je ne Je ne reviendrai pas sur les sondages, les pétitions, les mobilisations ou les délibérations prises en conseil municipal. Toutes ces actions ont conduit à construire et à réitérer le désir d'Alsace. Des milliers d'Alsaciens se sont exprimés. À cet appel, nous devons répondre par une action construite, institutionnelle et efficiente dans les domaines qui ont été déclinés dans l'accord de Matignon. À cet instant, je veux remercier tout particulièrement Mme la rapporteur, Agnès Canayer, de son écoute, de sa grande disponibilité et de son souci permanent d'accompagner ce texte jusqu'à la fin du parcours législatif dans les meilleures conditions possible. Je la remercie également d'avoir repris à son compte quelques-uns de mes amendements. Le texte Le texte de loi est un premier pas dans la bonne direction. Mais il ne va évidemment pas assez loin. Les coopérations transfrontalières doivent être renforcées. Je proposerai donc un amendement tendant à ce que la collectivité soit chargée d'organiser les modalités de mise en oeuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière. En matière de mobilité, l'Alsace doit pouvoir se battre à armes égales avec l'Allemagne contre le trafic insupportable des poids lourds, notamment en instaurant des contributions spécifiques qui pèseront sur les usagers des routes concernées. De plus, le texte doit prévoir la prise en charge par l'État des éventuels surcoûts des opérations de travaux inscrites au contrat de plan État-région 2015-2020 et transférées à la collectivité en 2021. du tourisme, de nouvelles prérogatives sont nécessaires. Je pense notamment à la possibilité donnée à la collectivité de coordonner sur son territoire la politique du tourisme. Enfin, si deux collectivités vont fusionner pour devenir une collectivité unique, originale, il n'est nullement question de fusion des deux entités administratives, même si le Gouvernement a exprimé un engagement en ce sens. Je vous présenterai donc un amendement à conforter la pérennité de la préfecture du Haut-Rhin comme chef-lieu de la nouvelle collectivité. Je vous rappelle qu'il en fut de même pour la région Grand Est et Strasbourg ; personne ne s'en est ému. Mon

Madame la présidente, madame le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi un instant de revenir en 2013. Nous proposions alors de créer une vraie région Alsace, regroupant les compétences de la région et des deux départements, avec des conseillers territoriaux pour élus. persuadé, la meilleure formule pour notre territoire et pour bien d'autres. Malheureusement, le référendum ne fut pas concluant. Ce fut pour moi un échec douloureux Mais rien n'étant jamais définitif, l'espoir revint le 22 janvier 2018, par le biais de la lettre de mission du Premier ministre demandant au préfet, M. Jean-Luc Marx, de mener une réflexion sur l'évolution des deux départements alsaciens.

Depuis la création, au 1 janvier 2016, de la région Grand Est, il n'existe plus de collectivité territoriale d'Alsace. » Troisièmement : « Au-delà des interrogations sur l'avenir administratif du territoire, le " désir d'Alsace " dépasse le registre institutionnel.

madame la ministre, lorsque, à la suite de ce rapport, vous avez organisé, avec vos services, de multiples réunions, aussi bien dans votre ministère qu'à l'occasion de nombreux déplacements en Alsace, ce dont je vous sais gré ! Vous connaissez par ailleurs la sympathie que je vous porte depuis bien longtemps. Espoir enfin, lorsque vous annonciez la volonté du Gouvernement de conclure cette démarche par une déclaration commune suivie d'un projet de loi. Mais l'espoir a rapidement cédé la place au doute le 29 octobre 2018, à la lecture de la déclaration de Matignon, que j'ai qualifiée le soir même, de « légère, voire transparente » ; elle reporte l'essentiel en 2021.

Oui, déception quant à la notion de chef de file à propos de l'action transfrontalière. Vous la bridez par de nombreux critères, à tel point que la nouvelle collectivité organisera peut-être, mais n'aura aucune compétence à décider. Gérer les fonds européens, par exemple, eût été une réelle compétence à lui confier. Déception encore, en constatant que le seul et réel transfert de compétence proposé est en réalité un transfert de charge à moyen et long termes. Je veux parler des routes nationales et des autoroutes non concédées. La charge nette est d'au moins 50 millions d'euros, compensation déduite. Belle opération de générosité de l'État à son propre égard

Déception enfin de constater que trop de mesures seront prises par voie d'ordonnance, alors qu'elles pourraient être utilement précisées dans la loi. Madame la ministre, j'ai salué votre qualité d'écoute. Je vous exhorte à entendre pareillement la demande des Alsaciens

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues,

qui seront peut-être utiles pour d'autres départements frontaliers, nous aurons réussi. Ayons donc ce débat sur la décentralisation au lieu de nous battre sur un nom qui va tromper les Alsaciens ; je pense qu'il faut leur dire la vérité. Ce que nous avons réussi est un pas, un petit pas. Mais le grand pas que nous devons à tous les Français, c'est une vraie décentralisation ; celle-là, nous ne l'avons pas !

Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, autant être clair tout de suite : la Collectivité européenne d'Alsace est une mauvaise réponse à une bonne et vraie question. Car même si ce projet de loi est censé mettre en oeuvre la déclaration de Matignon du 29 octobre dernier, les Alsaciens, dans leur immense majorité, n'ont jamais demandé la nouvelle structure territoriale qu'on leur propose Ils ont dit ce qu'ils revendiquent dans trois sondages successifs réalisés sur les deux dernières années, à savoir, pour plus de 83 % d'entre eux,

dès l'origine, ils ont fait partie de ces Français qui n'ont pas accepté le découpage totalement arbitraire et absurde des nouvelles régions, ainsi que la loi NOTRe qui a suivi. Leur souhait à ce jour reste le même revenir à la raison, grâce au retour à des collectivités régionales qui ont un sens en termes d'identité, d'espace et de projet. Ce serait pour eux, ce serait pour nous, ouvrir un nouvel acte de la décentralisation dans notre beau pays, la France Aujourd'hui, on leur propose de fusionner leurs deux départements en un, avec les seules compétences départementales, auxquelles on ajoute un unique transfert de la part de l'État, celui des routes non concédées et des autoroutes situées en Alsace. Autant dire que cette proposition ne les satisfait pas : ils entendent à tout le moins que d'autres compétences significatives soient ajoutées. Ce sera l'objet d'amendements qui vont être examinés tout à l'heure. Ce qui est au moins aussi grave, c'est que malheureusement ce texte suscite des incompréhensions dans les deux autres anciennes régions du Grand Est, en premier lieu chez nos collègues et amis de ces territoires, et qu'il divise, au lieu de rassembler sur les objectifs d'une vraie décentralisation que nous sommes nombreux dans cet voeux., il ne satisfait personne ! Sans compter que sur le plan juridique, le projet de loi soulève un certain nombre de questions que le Conseil d'État n'a pas manqué de relever, mais que le Gouvernement a décidé d'ignorer. La Haute Assemblée peut-elle sortir de ce débat par le haut ? À mon sens, oui, si elle voit dans la satisfaction du désir profond des Alsaciens une sorte de galop d'essai d'un acte III de la décentralisation pour notre pays. Il faut faire droit, mes chers collègues, à divers amendements déposés par les sénateurs d'Alsace, le premier d'entre eux visant à la reconnaissance dans cette Collectivité européenne d'Alsace d'une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution. Dès lors que ce statut lui aura été reconnu, des compétences spécifiques à son territoire, même si elles ne devaient s'exercer qu'à titre de chef de file, peuvent et pourront lui être dévolues. Ce serait un signe fort manifesté par le Sénat en faveur de la respiration de nos territoires. Cela pourrait incontestablement inspirer d'autres expériences dans notre pays.

La réforme mettant en place le conseiller territorial conservait la proximité avec l'élection cantonale, simplifiait et faisait économiser en supprimant les doublons entre le département et la région. Elle respectait la subsidiarité en permettant d'exercer chaque compétence à l'échelon le plus pertinent.

et reprendre l'idée du conseiller territorial. Il a décidé de maintenir ces grandes régions. Il est vrai que tous sont fatigués des réformes de structure, de l'intercommunalité à la région. la région. Elles accaparent les élus au détriment de leur mission, qui est d'abord de s'occuper des problèmes des citoyens et de soutenir des projets concrets. Or, quand on est accaparé par soi-même, on n'a pas le temps de s'occuper des autres. Mais ces grandes régions ne pourraient avoir un sens qu'avec des compétences et des moyens.

Ces grandes régions ne pourraient avoir un sens que par le transfert massif des compétences non régaliennes de l'État, avec les moyens correspondants. Mais voilà, l'État ne lâche pas prise. L'État, qui est en difficulté, pour ne pas dire en faillite, quant à ses missions régaliennes, si l'on en juge par l'état matériel des armées et de nos forces de sécurité intérieure, et pire encore de la justice- juridictions et administration pénitentiaire -, aurait tout à gagner à se concentrer sur le régalien.

Or il cherche toujours à régenter la mise en oeuvre des compétences décentralisées. Il n'y a plus de doublons entre les collectivités territoriales, mais il y a systématiquement doublon entre l'État et les collectivités.

de la technostructure d'État, et ce, à la lettre. pour les régions en matière de formation. L'État devrait aussi et surtout transférer ses compétences non régaliennes aux régions : le service public de l'emploi, celui de l'orientation, l'environnement, les routes

des territoires de notre pays. Au-delà de la question juridique et constitutionnelle, j'ai également expliqué comment une solution acceptée pour une collectivité, mais refusée pour sa voisine,

Pour autant, je ne crois pas que le régime concordataire ait beaucoup de rapport avec les compétences dont nous parlons ce soir, je pense notamment à la gestion des réseaux autoroutiers et à la promotion du bilinguisme

Nous nous trouvons dans une situation qui est acquise : la fusion existe ; elle a été acceptée par les présidents des conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, et par le président du conseil régional ; le décret a été pris tous les accords ont été négociés avec l'État. Nous sommes aujourd'hui en situation de discuter des compétences, nous sommes aussi en situation- ce point n'a pas été évoqué, car il fait consensus -de discuter de la migration des personnels et des moyens du transfert des compétences. C'est ici et maintenant qu'il faut le faire,

Mais ce n'est pas le sujet ce soir. Ce soir, prenons le temps de discuter de ce projet de loi dont le manque d'ambition a été relevé par nombre d'entre nous. Prenons le temps de l'améliorer. Prenons le temps d'offrir aux Alsaciens

Bas-Rhin. Cet amendement vise à mettre en oeuvre une consultation des électeurs du département d'Alsace, d'Alsace, qui, dans une logique de référendum local, a pour objet de demander aux Alsaciens s'ils souhaitent ou non le rétablissement d'une région d'Alsace de plein exercice.

amendements, puisqu'ils visent à recourir au référendum pour la sortie de l'Alsace du Grand Est- soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la loi -alors même que le département d'Alsace n'existe pas encore.

une situation transfrontalière avec pour voisins des collectivités dotées d'une grande autonomie, le dynamisme d'une langue et d'une culture qui façonnent leur caractère particulier. particulier. La création d'un département unique d'Alsace est nécessaire, tant la refonte de la carte régionale a balayé d'un revers de main l'histoire et la géographie et a donné naissance à des ensembles monstrueux sans identité. Ah ça ! Comment imaginer que l'Alsace, rayée d'un trait de plume, n'allait pas réagir ?

À défaut, donnons au moins à ce département unique d'Alsace de réelles compétences en matière d'éducation, de politique linguistique, de culture, de mobilité ou de gestion transfrontalière, faute de quoi nous créerions un ersatz et beaucoup de désillusions. Le Sénat étant la chambre des territoires, répondons à leurs attentes ! Nous le savons, ils ont besoin de liberté et certains d'entre eux, qui doivent affronter des questions spécifiques, d'un statut particulier, qui n'altérera en rien leur intégration dans la communauté nationale et dans la République.

D'une part, il se limitait à ériger la désormais disparue Collectivité européenne d'Alsace en chef de file de la coopération transfrontalière sur son territoire, en maintenant les pouvoirs de l'État et de toutes les autres collectivités. D'autre part, en matière de langue et de culture régionales, il se contentait de faire référence à la convention quadripartite d'ores et déjà signée, pour la quatrième fois, entre l'État, la région et les deux départements du Rhin. Fort heureusement, toutefois, la commission des lois a commencé à lui donner un peu de contenu en adoptant des amendements portant sur la formation des enseignants en langue et culture régionales, sur l'ouverture de classes bilingues et sur la promotion de la langue régionale. Il convient désormais, mes chers collègues, d'aller plus loin et d'inscrire dans ce texte que la collectivité territoriale dont il est question est une collectivité à statut particulier au titre de l'article 72 de la Constitution.

Je considère en particulier inacceptable que l'amendement n° 100, qui tendait à ce que la collectivité à statut particulier dispose des compétences des régions, ne puisse pas être discuté, sous le prétexte qu'il serait irrecevable au titre de l'article 40. Je suis d'autant plus surpris que j'avais déposé le même amendement

quand on élabore une législation spécifique à une région, il est préférable de rappeler rapidement son histoire. Dans le cas de l'Alsace, cela permet de comprendre son particularisme et son attachement à l'Europe. La plupart des régions frontalières de notre pays ont une histoire douloureuse, mais cela est particulièrement vrai pour l'Alsace depuis la désastreuse guerre de 1870. Malgré la « protestation solennelle de Bordeaux » élevée par ses députés, l'Alsace-Moselle a été cédée au nouvel empire allemand. De la protestation, l'Alsace est passée à la résignation puis à l'autonomisme, en réaction à la politique de germanisation. Lors de la Première Guerre mondiale, des membres d'une même famille se sont trouvés dans les deux armées ennemies. Après le retour à la France, l'Alsace a connu le clivage entre les autonomistes et les nationalistes, entre la défense du particularisme et la résistance au jacobinisme parisien. L'étrange défaite de 1940 a permis à l'Allemagne d'annexer de nouveau l'Alsace et la Moselle. Les nazis y menèrent propagande et répression, imposant l'obligation de germaniser les noms et les prénoms. C'est surtout la tragédie de l'incorporation de force dans l'armée allemande qui a marqué durablement la psychologie alsacienne, avec 42 000 morts ou disparus sous l'uniforme allemand.

Pierre Pflimlin a été le chantre inlassable de l'Europe et de la vocation européenne de Strasbourg, symbole de la réconciliation et de l'amitié entre la France et l'Allemagne. C'est ainsi que Strasbourg est devenue le siège du Conseil de l'Europe, de la Cour européenne des droits de l'homme, du Parlement européen et de la chaîne Arte. Cet ancrage de l'Alsace dans l'Europe lui a permis de sauver le référendum de François Mitterrand sur le traité de Maastricht en 1992. À l'histoire s'ajoutent deux réalités quotidiennes chaque jour, 25 500 frontaliers vont travailler en Allemagne, et 33 200 en Suisse alémanique ; notre langue régionale s'exprime par écrit en allemand standard et oralement par des dialectes. Il en résulte une coopération transfrontalière ancienne et intense. Le vocable « européen », sur lequel nous aurons à nous prononcer tout à l'heure, est donc pour l'Alsace non pas une incantation, mais une réalité vécue, voire une nécessité.

en présence de l'ensemble des parlementaires des deux départements. C'est un projet « cousu main », avez-vous alors indiqué, madame la ministre.

Le Sénat, chambre des territoires, se doit d'être un moteur et un facilitateur de ce premier pas, de ce premier exemple, qui se trouve être alsacien.

l'Alsace et le sujet qui nous occupe, vous déclarez : « ces nouvelles attributions préfigurent [ ...] le principe de différenciation des compétences des collectivités territoriales qui a été proposé par le Gouvernement dans le cadre de la révision constitutionnelle. Mes chers collègues, Mme Gourault nous emmène sur un tout autre terrain que la question du « désir d'Alsace » : il s'agit de la révision constitutionnelle

rétropédalage sur certains aspects et désaccord sur d'autres, nous avons adopté des ajustements sur la question de l'eau et de l'assainissement, notamment, à l'unanimité.

il n'est pas au rendez-vous des territoires ni au rendez-vous des responsabilités ! Vous faites fausse route. Levez le crayon, il n'est pas trop tard ! Laissez un peu de temps au grand débat et offrez à la représentation nationale, ainsi qu'à l'ensemble des élus des territoires, un moment de répit

ont souhaité que les deux départements fusionnent pour former une seule collectivité, la Collectivité européenne d'Alsace.

Masson. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues,

Et je ne pense pas que nous vous demanderons à l'avenir l'autorisation de continuer de le faire ! Le véritable problème auquel nous sommes confrontés, c'est l'asymétrie complète des compétences. Pour pouvoir aller discuter avec le président du gouvernement autonome basque ou le président de la communauté autonome de Navarre,

Ainsi, le projet de loi reconnaît à la nouvelle collectivité un rôle de chef de file en matière transfrontalière, en particulier l'élaboration d'un schéma de coopération transfrontalière, lequel schéma comportera un volet opérationnel, y compris pour les liaisons routières et ferroviaires. ferroviaires. Il lui reconnaît également un rôle renforcé en matière de langue régionale, dont je rappelle que son expression écrite est l'allemand standard. La dénomination de la nouvelle collectivité européenne exprime donc son ambition transfrontalière et renforce sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires allemands et suisses. Deuxièmement, malgré cette volonté politique forte, votre commission des lois a préféré suivre prudemment l'avis du Conseil d'État, qui a opté pour la dénomination « département d'Alsace ». Toutefois, deux observations s'imposent : tout le Conseil d'État a validé l'attribution des compétences spéciales de la nouvelle collectivité, reconnaissant ainsi la spécificité de l'Alsace ;

Toujours sur le plan juridique, je ferai observer que le décret du 27 février 2019 a procédé au regroupement des deux départements rhénans sous le nom de Collectivité européenne d'Alsace. en application de l'article L. 3111-1 du code général des collectivités territoriales, seul un nouveau décret pris sur demande de la nouvelle collectivité peut modifier cette dénomination. Troisièmement- l'argument est très politique, j'en conviens -, la dénomination « Collectivité européenne d'Alsace » permettra une identification forte par les Alsaciens et, par là même, mettra du baume au coeur des 85 % d'Alsaciens qui ne veulent pas rester des « Grands Estiens

par trois fois : dans la déclaration commune du 29 octobre 2018, dans les délibérations des deux assemblées départementales adoptées le 4 février 2019 et dans le décret du 27 février 2019 ayant procédé à la fusion des départements. La dénomination de la collectivité relève, à mon sens, du domaine réglementaire, et la question a été traitée par décret. Revenir par la loi sur ce point ne me paraît pas judicieux. Par ailleurs, l'attente des Alsaciens et le contenu même du projet plaident pour conserver le nom choisi.

chef de filât en matière transfrontalière, rôle renforcé dans la promotion des langues régionales. Mes chers collègues, le nom « département d'Alsace » ne serait pas conforme à la réalité territoriale et institutionnelle nouvelle. si la future collectivité se résumait à un département d'Alsace, il n'y aurait pas besoin de loi, et nous ne serions pas ici ce soir ! L'appellation « Collectivité européenne d'Alsace »,

Enfin, comme je le rappelais lors de la discussion générale, l'attente alsacienne sur ce point est grande et l'identification avec cette dénomination est forte. Le désir d'Alsace ne peut être réduit à un désir de département ! Pour l'ensemble de ces raisons, mes chers collègues, je vous demande de rétablir le nom que

un département doté de nouvelles compétences, mais c'est un département avant tout ! Le terme « Collectivité européenne d'Alsace » est un nom propre et, à

décision a été prise à la majorité absolue du conseil départemental du Haut-Rhin

« le respect des compétences des autres catégories de collectivités territoriales ou de leurs groupements », mais ayons le courage de le dire : « Ça suffit ! » Après avoir prévu que le schéma transfrontalier doit être en

et sa strate de rattachement sont deux sujets qu'il faut bien dissocier. La parole est à M. Jacques Bigot,

un terme plus flatteur, plus séduisant, plus vendeur, mais aux mots qui flattent, je préfère ceux qui disent la vérité de ce qu'ils recouvrent.

si le Gouvernement a vraiment une opinion. C'est

il faut, pour faire un pâté aux alouettes, un cheval et une alouette. Nous avons là un département, qui n'est pas simplement un département : c'est un département plus quelque chose.

La chose, c'est un département créé par décret. Celui-ci n'a nul besoin d'une loi pour voir le jour. Et si le Gouvernement a estimé qu'il fallait une loi, c'est que, en réalité, nous sommes en train de créer un peu plus

C'est ainsi que, au-delà des compétences que le Gouvernement avait prévues, notamment en matière routière ou transfrontalière, nous avons ajouté la promotion de l'attractivité, qui était une compétence jusque-là réservée à la région, nous avons ajouté la qualité de chef de file en matière de bilinguisme, et nous nous nous nous apprêtons à ajouter la coordination de la politique touristique, l'expérimentation des aides aux entreprises par délégation de la région, des pouvoirs de police

Nous proposons également la création d'un conseil de développement, ainsi que la possibilité de créer dans ce département particulier une télévision locale, pour défendre la langue alsacienne. Je comprends que dans la perspective ouverte par le Gouvernement, qui a désiré faire plus qu'un département, le Sénat s'apprête à faire beaucoup plus qu'un département, sans pour autant créer une collectivité à statut particulier. Eh bien, mes chers collègues, vous connaissez la position de la commission, mais, en votre âme et conscience, vous allez pouvoir maintenant dire si vous souhaitez que l'on s'en tienne à la dénomination « département », ou si, tenant compte de toutes ces avancées, vous préférez aller plus loin. Peut-être choisirez-vous alors de reprendre la dénomination qu'ont retenue tant les conseils départementaux d'Alsace que la région Alsace, ainsi d'ailleurs que le Gouvernement. Cela, c'est votre appréciation. Je le rappelle encore une fois, la position de la commission était différente.

pour créer une collectivité dotée de compétences particulières et supplémentaires. » N'est-ce pas la définition même d'une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution ? Pour moi, cette collectivité, c'est un espace, c'est une identité, c'est un projet. Par Par ailleurs, le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, a clairement indiqué que la Collectivité européenne d'Alsace, créée par décret, n'était en fait qu'un département auquel il avait été ajouté des compétences d'intérêt général spécifiques à ce territoire.

à ce que prévoit déjà le projet de loi, même s'il tend à autoriser ultérieurement le législateur à attribuer d'autres compétences à la collectivité alsacienne, sans qu'il soit besoin de le justifier par des spécificités locales. locales. Il me semble que cette solution hybride poserait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait. D'un point de vue politique, il faudrait toujours justifier les compétences spéciales de la collectivité alsacienne par des spécificités locales, faute de quoi les autres territoires de la région ne le comprendraient pas. En outre, si l'on en venait à attribuer à la collectivité des compétences aujourd'hui exercées par la région, il en résulterait que la région Grand Est exercerait depuis Strasbourg, sur le territoire de la Moselle ou de la Marne, des compétences qu'elle n'aurait même pas le droit d'exercer en Alsace.

quelques compétences supplémentaires au regard de sa situation spécifique. Madame la ministre, je me suis certainement mal fait comprendre, car j'avais le sentiment d'avoir démontré l'inverse, à savoir qu'il ne pouvait s'agir, juridiquement, que d'une collectivité à statut particulier ! Je le

l'on applique la jurisprudence du Conseil d'État sur l'affectation de compétences nouvelles à une strate de collectivités locales, il est clair que cela ne peut plus être un département.

il nous a finalement invités à choisir le nom de Collectivité européenne d'Alsace. En outre, il a recensé toutes les compétences

qu'il m'est arrivé, dans d'autres territoires, de manifester en faveur d'une collectivité à statut particulier. De surcroît, c'est la réalité de ce que nous allons constituer, puisque nous allons donner à ce « département + » un certain nombre de compétences tout à fait spécifiques.

s'agissait d'un département avec quelques compétences supplémentaires, mais globalement accessoires, que l'on ne devait pas l'appeler « département », bien que c'en était un, et qu'un nom unique, propre, allait qualifier cette Collectivité européenne d'Alsace.

pas ? Nous voulons appliquer par la loi l'accord qui a été signé entre la région, les deux départements et le Gouvernement. C'est aussi simple que cela. Par ailleurs, fondamentalement, la Collectivité européenne d'Alsace fait partie de la catégorie des départements,

bien, les collectivités à statut particulier sont des collectivités qui ont deux couches, si je puis dire, de collectivités territoriales.